cet amendement pénaliserait donc les contribuables concernés plutôt que de les aider. En revanche, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, si la cotisation obligatoire de sécurité sociale est précomptée au dû, au titre de revenu exonéré, elle ne peut pas être déduite du montant des autres revenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu. En tout état de cause,

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 du code général des impôts. Serait ainsi assurée l'application uniforme du prélèvement forfaitaire unique à 30 % instauré par la loi de finances pour 2018, quelle que soit l'étendue de l'assiette d'imposition. L'objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d'imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d'imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

dans des circonstances pénibles, les droits de succession viennent s'ajouter à une longue chaîne de taxation des revenus de l'épargne, selon des tarifs souvent fortement progressifs. Cet amendement, présenté par l'ensemble des membres de notre groupe, vise à resserrer l'assiette des droits de succession en transformant l'abattement de 20 % actuellement prévu sur la valeur de la résidence principale en un abattement de 600 000 euros.

cet amendement permettrait donc d'exonérer de droits de succession un nombre significatif de résidences principales, tout en maintenant l'application de ces droits pour les contribuables les plus fortunés. Quel

Un tel délai n'était pas requis avant 2006. Fixé ensuite à six ans, il a progressivement été relevé à dix ans, puis à quinze ans. L'abaisser à huit ans permettrait de revenir à un délai plus raisonnable et plus respectueux des droits des contribuables.

Aussi, je propose de porter à 100 000 euros l'abattement s'imputant sur la valeur des dons d'argent réalisés au profit des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, et de réduire à dix ans le délai à respecter avant de pouvoir réitérer un don dans les mêmes termes.

donations, soit un niveau d'imposition deux fois plus élevé qu'au Royaume-Uni et trois fois plus important qu'en Allemagne. Il s'agit là d'une fiscalité que les Français perçoivent à juste titre comme confiscatoire. L'objet de cet amendement est de porter de 100 000 euros à 200 000 euros l'abattement s'imputant sur la valeur de la part de chaque héritier.

François Bonhomme. Cet amendement vise à favoriser la transmission entre générations en permettant aux grands-parents de donner à leurs petits-enfants, avant que ceux-ci n'aient atteint l'âge de trente ans, des parts de capital, à condition que leur usufruit soit transféré à des associations reconnues d'utilité publique ou à des fondations. Dans cette hypothèse, cet amendement vise à exonérer une telle donation de droits de mutation.

à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs, il n'y aurait pas d'effet pédagogique pour celui qui reçoit, dans la mesure où il est mineur, donc, par définition, extrêmement jeune. En outre, l'aide au démarrage dans la vie active ou dans la vie d'adulte serait empêchée par le délai minimum de dix ans

Cet amendement vise à éviter que les plus-values sur titres, qui font depuis le 1 janvier 2018 l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique au titre de l'impôt sur le revenu et et des prélèvements sociaux- disposition tout de même assez unique en Europe ... -, soient en sus soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, actuellement due en application des dispositions des articles 223 et 1417 du CGI. L'objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d'imposition des investissements en capital. Son adoption confirmerait la volonté du législateur de rapprocher le taux français d'imposition des plus-values sur titres des taux en vigueur chez nos voisins européens.

1771 et qui concerne le salaire du conservateur des hypothèques. Le conservateur des hypothèques n'existe plus. Pourtant, son salaire existe toujours ! Cela signifie en clair que, quand un créancier

dont une partie concerne le salaire du conservateur des hypothèques, qui n'existe plus depuis l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010. L'objet de cet amendement est extrêmement simple : le conservateur des hypothèques n'existant plus, il serait logique et bienvenu de supprimer le salaire

le retire, monsieur le président que 5,5 % de l'épargne salariale aujourd'hui en France. À cet effet, il est proposé d'étendre la mesure d'exonération du forfait fiscal de 20 % à l'ensemble des flux d'épargne salariale investis dans des fonds solidaires. Il est assez paradoxal, pour ne pas dire plus, que l'État prélève 20 %, au titre d'un forfait dit « social », des sommes investies sur une durée de cinq ans par les salariés dans un but de solidarité et d'utilité sociale. En élargissant l'exonération du forfait social aux fonds solidaires, le Gouvernement donnera un signal de mise en oeuvre concrète de la stratégie. Quel est l'avis

Décision a été prise de verser au fonds spécifique qui accompagne les rénovations du patrimoine une somme supplémentaire de 21 millions d'euros en plus des gains liés aux seuls achats de tickets du loto du patrimoine.

cette année, mais qu'en sera-t-il l'année prochaine et la suivante ? En faisant figurer dans la loi une modalité précisant que l'État ne perçoit plus la taxe, mais que c'est le jeu lui-même qui finance

Quand il n'y a plus de réserve parlementaire, ... Ah oui ! ... quand toutes les dotations des territoires et des collectivités sont en chute libre et quand les budgets sociaux des départements l'emportent sur l'entretien du patrimoine, un tel jeu n'est ni un luxe

Je suis la présidente de l'Association Petites cités de caractère de France, qui compte plus de 160 communes. La plupart d'entre elles ont moins de 600 habitants. Leur seul levier d'avenir, c'est leur patrimoine, qui est générateur d'une économie touristique non négligeable. Quand des citoyens s'engagent pour aider l'État

On ne peut pas confondre ce type de loto avec les autres jeux. C'est le Président de la République lui-même qui en a fait une cause nationale et qui a invité chaque Français à contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Soutenons les très bons citoyens

contributions étaient en partie destinées à amortir les effets de la condamnation de notre pays pour l'imposition exceptionnelle des dividendes. Nous, nous disons : vive l'impôt ! À condition qu'il soit juste, équitable, progressif, et surtout que personne n'y échappe.

les structures spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l'écoute et l'orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes. répond en partie à l'appel de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, pionnière en la matière, qui milite pour la multiplication de telles structures.

le nécessaire développement de structures d'accueil médico-sociales des victimes de violences sexuelles ou sexistes. Cet amendement tend à créer un cadre juridique adapté et

l'avis du Gouvernement ? Je confirme l'analyse de M. le rapporteur général. Selon l'article 200 du code général des impôts, le fait d'avoir une gestion désintéressée, d'être à but non lucratif et de ne pas agir pour un cercle restreint de personnes ouvre droit au mécénat.

qui font du mécénat. Je le répète, si les très grandes entreprises financent le mécénat culturel à hauteur de 70 %, les petites et moyennes entreprises y concourent trop peu, en raison notamment des dispositions qui limitent le bénéfice de la réduction fiscale aux versements inférieurs à 0,5 % du chiffre d'affaires des entreprises. Cet amendement tend donc à étendre, comme l'a dit le rapporteur général, le bénéfice de la réduction fiscale aux dons annuels inférieurs à 10 000 euros, y compris lorsqu'ils excèdent 0,5 % du chiffre d'affaires des entreprises mécènes.

PME ont beaucoup insisté sur le lien entre le territoire et leur entreprise. Pour eux, le mécénat est un vecteur

La gouvernance des SPL est publique à 100 %. L'actionnariat de ces sociétés est composé exclusivement des collectivités publiques, lesquelles exercent sur la SPL un contrôle analogue à celui que celle-ci exerce sur leurs services. La souplesse de gestion de la SPL en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, notamment pour le service public culturel. et de la répression des fraudes, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les SPL, entités distinctes, mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également l'une de leurs principales qualités, les SPL faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France, par l'État, les chambres régionales des comptes, les commissaires aux comptes, les collectivités actionnaires, etc. Les SPL, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en oeuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d'égalité avec les autres acteurs publics, alors qu'elles ont pour objet la gestion d'un service public. Cela pénalise leur activité. Pourtant, l'article 238 du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l'État en est actionnaire. reconnaître la possibilité d'un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 21 septembre dernier. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les SPL, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal C'est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, vise à proposer une évolution de l'article 238 du code général des impôts, afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat. Les collectivités territoriales jouent aujourd'hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d'équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés, afin de faire face à la baisse des dotations de l'État.

aux sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales. En effet, de nombreuses collectivités font aujourd'hui le choix de confier à des sociétés publiques locales des missions d'intérêt général, notamment la gestion d'équipements culturels

Lavarde. Cet amendement tend à élargir au domaine sportif des dispositions s'appliquant dans le domaine de la culture, notamment permettre la prise en charge de certains frais d'organisation d'une manifestation à but caritatif par des entreprises dans le cadre du mécénat. Cela permettrait d'améliorer le bénéfice reversé à la cause soutenue. Nous estimons que ce qui peut s'appliquer au spectacle vivant peut aussi s'appliquer au spectacle sportif.

versante aux dons effectués dans le cadre de l'accompagnement du double projet d'un sportif de haut niveau. Cette disposition existe d'ores et déjà dans le mécénat culturel. En effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d'associer son identité à celle de l'artiste qu'elle souhaite soutenir au travers d'une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif. Il importe de souligner ici que cette démarche se différencie du, puisque la fondation dispose d'un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formation. Le dispositif proposé ici s'adresse à des sportifs peu connus ou inconnus du grand public, qui représentent l'avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s'inscrire dans une démarche de commercial.

quand le don est à destination du sport pour les personnes handicapées ou du développement de la pratique du sport adapté. Aujourd'hui, ce sont trop souvent des opérations de ou des manifestations qui viennent soutenir les athlètes handisports.

lui affectant irrévocablement ses versements ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % des versements, ce qui est déjà un dispositif très attractif et généreux pour assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine. Les monuments historiques bénéficient

actions, après la suppression de l'ISF-PME, il ne restera plus de différence majeure, sauf un Madelin plafonné dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine, entre la fiscalité qui s'applique aux produits d'un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s'applique aux produits des premiers investissements dans les start-up, qui, chacun le sait, ont besoin d'une forte capitalisation au départ pour réussir.

régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines de la nouvelle économie. Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux vers leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s'imputent sur le revenu imposable de l'actionnaire et ne sont plus reportables pour l'entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l'investissement. En régime de croisière, l'IS des ayant réussi représente trois fois la perte d'IR due à l'imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué. L'idée est donc de reprendre en France ce dispositif qui existe aux États-Unis. Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur le sujet.

Pour mémoire, le régime de l'article 239 AB du code général des impôts déroge au régime du droit commun des sociétés de capitaux, qui relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés. Cet article permet à la société, pourvu qu'elle soit constituée d'au moins 50 % d'associés personnes physiques, d'opter pendant cinq exercices pour l'application de l'impôt sur le revenu. Votre proposition consistant à limiter l'application de l'impôt sur le revenu au montant de l'investissement en capital des associés impliquerait de liquider, pour un investisseur donné, le bénéfice imposable, à la fois selon les règles de l'impôt sur les sociétés et selon les règles de l'impôt sur le revenu. Il y aurait donc deux dispositifs fiscaux pour un même associé, ce qui nous paraît constituer une source de complexité. une source de complexité. En outre, l'enjeu de l'instauration de ce dispositif optionnel en 2008 avec la loi de modernisation de l'économie était de permettre aux associés professionnels personnellement impliqués dans le développement de l'entreprise d'imputer les déficits des premières années d'activité sur leur revenu global, ce qui rejoint l'amendement de M. Cadic. Les règles déterminant quels associés sont considérés comme professionnels n'ayant pas été modifiées, les associés passifs qui se contentent d'apporter des capitaux dans la société ne bénéficient pas de ce régime pour le déficit leur revenant. Or votre proposition va plus loin en permettant à tout associé, qu'il soit actif ou passif dans la société, d'imputer sur son revenu global la quote-part des déficits lui revenant à hauteur de son investissement. Enfin, le régime de l'article 239 AB du code général des impôts est réservé aux sociétés dont les dirigeants détiennent au moins 34 % du capital. Il a pour but de réserver l'application du régime aux sociétés dont les dirigeants s'impliquent personnellement sur le plan financier et conservent une minorité de blocage leur permettant de s'opposer à des décisions leur paraissant contraires à l'intérêt de la société. Il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce principe de gouvernance des entreprises concernées. Pour ces trois raisons- la complexité

n° I-106 rectifié. L'article 18 du projet de loi de finances pour 2019 porte sur la réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles, fruit des travaux du groupe de travail réunissant l'ensemble des acteurs du secteur, les organisations syndicales, les professionnels agricoles, ainsi que les parlementaires. Nous avons oeuvré, tous ensemble, pour essayer de trouver des avantages à cette profession. Force est de constater que la capacité d'épargne des entreprises agricoles varie selon les années, en raison notamment de l'investissement, de l'activité ou de sa taille. Le résultat d'exploitation traduit par le plan comptable agricole donne une parfaite vision de la performance économique annuelle et de la capacité à épargner de l'entreprise agricole, alors que le résultat fiscal n'est pas nécessairement directement connecté à la capacité d'épargne, générant des retraitements fiscaux complexes pour déterminer l'assiette fiscale. En se fondant sur une assiette fiscale comme le chiffre d'affaires, on risque de voir le dispositif d'épargne de précaution tomber sous la règle, règlement mis en place par l'Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises, le dispositif pouvant être requalifié comme une forme d'aide d'État de nature fiscale et perdant en efficacité. Par conséquent, le présent amendement vise à substituer un indicateur comptable, le résultat d'exploitation, à l'assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.

je propose de substituer un indicateur comptable, en l'occurrence le résultat d'exploitation, à l'assiette fiscale. On ne peut pas se fonder sur une assiette fiscale comme le chiffre d'affaires, car cela ferait tomber le dispositif d'épargne de précaution sous le coup de la fameuse règle, comme l'a rappelé Daniel Laurent. En effet, le mécanisme pourrait alors être considéré comme une sorte d'aide d'État de nature fiscale.

à opérer un complément de déduction en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen, et ce afin de prendre en compte la diversité des exploitations agricoles françaises et de leurs profils économiques.

qui, dans la rédaction actuelle de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2019, est propre à chaque contribuable. Afin de clarifier ce point et d'accroître la lisibilité de cette donnée fondamentale, il est proposé d'instituer la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre

La dispense d'épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle qu'elle est prévue par le texte issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, est concrètement inapplicable, particulièrement s'agissant de l'obligation de reconstitution de l'épargne monétaire lors de la vente desdits stocks. Comment imaginer, par exemple, qu'à chaque vente de bouteille, un viticulteur se doive de penser à créditer le compte épargne d'un montant au moins égal à la différence entre 50 du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ? Le présent amendement vise à permettre la dispense d'épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.

l'article 18, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation puisse se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant. prévoyons également que la déduction fiscale sera définitivement acquise si l'épargne monétaire est constituée dans un délai raisonnable, à la clôture du troisième exercice pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits agricoles, et maintenue jusqu'au terme du délai du dixième

restreindre la faculté de satisfaire de façon équivalente la condition d'épargne sous une forme monétaire ou réelle. En conséquence, la commission

fait partie des moyens permettant de gérer au mieux, notamment à partir des stocks, les aléas climatiques.

L'article 18 du projet de loi de finances pour 2019 permet la constitution d'une épargne pour encourager les exploitants agricoles à se prémunir individuellement contre les risques et les aléas.

pour investissement des acquisitions d'immobilisations amortissables. Le cumul de la nouvelle incitation fiscale à l'épargne de précaution et la non-imposition des plus-values issues de la cession de matériel relancent la surmécanisation dans les exploitations agricoles qui réalisent moins de 250 000 euros de recettes. Le délai de deux ans imposé entre la constitution de l'épargne et la revente correspond, sur le marché des matériels agricoles saisonniers, à une utilisation sur une seule campagne. Il est donc manifestement insuffisant. De plus, le montant de la plus-value sur deux ans est inférieur, selon les exemples pris en compte par les professionnels, à celui de la plus-value sur trois ans. Un délai plus important est donc indispensable pour prévenir des comportements de surinvestissement en matériel que pourrait susciter la déduction pour épargne de précaution.

Dans la vie, il peut se produire des cessations totales ou partielles d'activité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole.

Par exception, lorsque l'activité principale de la société civile est de nature agricole, les recettes accessoires de nature commerciale sont imposées comme des bénéfices agricoles, lorsque la moyenne des recettes tirées de l'ensemble des activités accessoires des trois années civiles précédentes n'excède ni 50 % de la moyenne du chiffre d'affaires agricole apprécié sur la même période, ni 100 000 euros. Sans avoir à se transformer en société commerciale, les sociétés civiles agricoles peuvent réaliser des activités non agricoles. Aussi, je crains que votre proposition ne soit dénuée de portée dans un certain nombre de cas. En adoptant une forme commerciale, les exploitants agricoles basculent presque toujours dans l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cette circonstance rendra inapplicable le mécanisme de dispense de réintégration. Cependant, le projet de loi de finances que nous vous présentons comporte deux nouveaux mécanismes encourageant les agriculteurs à opter pour l'impôt sur les sociétés, pour atténuer les conséquences liées au passage de l'impôt sur le

selon un régime réel d'imposition. Les sociétés exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution. Le présent Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante, soit avec un chiffre d'affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d'affaires global de la société. La parole est à M.

est l'objet de cet amendement.

constituerait une remise en cause du principe d'unicité de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, car les entreprises agricoles

Bel Maille est une entreprise installée à Riorges, près de Roanne, où l'industrie textile a un ancrage historique. Cette entreprise était européen de la création et de la fabrication de tissus en maille. suite du rachat de l'usine par un nouveau patron, qui s'identifiait comme entrepreneur, mais qui n'était pas là pour servir les intérêts de l'entreprise, Bel Maille s'est effondrée. Pendant des mois, ce sont les salariés qui se sont mobilisés pour défendre leur outil de travail et le savoir-faire d'excellence qui a été forgé année après année. Cet amendement a trois objets. Tout d'abord, en cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n'auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l'opération de cession. Le cessionnaire pourra donc, à ce titre, être condamné à rembourser les sommes perçues. Ensuite, est créé un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d'entreprises, visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l'instauration d'une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d'avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s'agit d'étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d'entreprises industrielles. Enfin, nous proposons la réévaluation du plafond d'exonération de l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d'une PME appartenant à une branche d'activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale,

À ce titre, le plafond d'exonération de l'impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes, et de vingt à trente points pour les petites entreprises, le tout sans toucher au plafond fixe de 7,5 millions d'euros.

à compter du 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2022, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible, par exemple un nouvel équipement industriel, de bénéficier d'un avantage fiscal exceptionnel, qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien. Cette mesure, qui a pris fin le 14 avril 2017, s'est révélée pleinement efficace, puisque l'investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d'euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d'euros entre 2016 et 2017. Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions et 800 millions d'euros par an.

Il tend également à mettre en oeuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la réforme de la fiscalité agricole. L'objectif est simple : sécuriser la constitution des sociétés agricoles, qui sont aujourd'hui un mode de regroupement privilégié, et l'un des moyens à disposition des exploitants agricoles pour renforcer leur compétitivité et faire face aux différents risques auxquels leur activité est soumise. Cet amendement tend

l'impôt sur les sociétés résulte d'un choix personnel de l'exploitant agricole. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire de transposer le régime de neutralité fiscale aux fusions de sociétés civiles agricoles, dès lors qu'il existe déjà des mécanismes atteignant les effets fiscaux de certaines transformations. En cohérence avec

au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et non au titre des bénéfices agricoles. Or ces activités, juridiquement agricoles, ne proviennent pas de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts. Plusieurs types d'activité ayant pour support l'exploitation sont concernés comme la restauration, la location de chambres d'hôtes au sein de l'exploitation ou encore le camping à la ferme. Or il n'est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle leur activité. Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l'exploitation. Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.

dans le revenu considéré comme agricole d'autres revenus sous réserve de respecter des plafonds, nous ne voyons pas d'autre objectif à ces amendements que de supprimer les plafonds et d'assujettir

Le coefficient multiplicateur était justifié par la différence de chiffre d'affaires entre les producteurs intégrés et ceux qui vendent leur production ; cette différence n'est plus constatée aujourd'hui. Or ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values. Cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est souvent le cas à cause du coefficient d'intégration. Les capacités d'investissement des producteurs de veaux s'en trouvent affectées. Il est donc proposé ici de réduire le coefficient multiplicateur de trois points, c'est-à-dire de le ramener à 2.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement de notre collègue Alain Bertrand a pour objet d'aligner le régime d'imposition des subventions et primes d'équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations. Quel

les entreprises de travaux agricoles dont le métier est de réaliser des travaux agricoles pour le compte d'exploitants agricoles. Cette problématique a été soulevée lors de l'examen du projet de loi sur l'agriculture. Le doublement des seuils prévus à l'article 75 du code général des impôts

L'article 18 précise seulement que les revenus tirés de l'exercice des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole mentionnées au premier alinéa de l'article 75 du CGI ne peuvent pas donner lieu à la déduction pour épargne de précaution. La réalisation d'activités accessoires à la production agricole est prise en compte pour faciliter la diversification des activités des exploitations agricoles : vente à la ferme, gîtes, chambres d'hôtes. Parmi ces recettes, figurent les recettes commerciales issues d'activités de travaux agricoles qui ne relèvent ni de l'entraide, de l'entraide, ni de l'échange, ni de l'achat collectif de matériels agricoles. Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles sont censés faciliter la diversification des activités

Il est donc proposé d'exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales visées à l'article 75 du code général des impôts.

pour 2018, afin de créer un régime unique applicable à l'ensemble des recettes accessoires perçues par les exploitants agricoles, qu'elles soient liées à la production d'énergie ou à d'autres activités.

et les parachutes dorés de complaisance, en taxant ces indemnités à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net.

effectué sur les entreprises non-résidentes ayant une activité économique numérique importante sur le territoire national. Le principe est simple : si une entreprise est simple : si une entreprise numérique a une activité suffisamment importante en France, ses revenus tirés de son activité française doivent être déclarés au fisc français. Elle devra alors payer l'impôt sur les sociétés sur ces revenus, au même titre que les autres entreprises exerçant sur le territoire national. Il s'agit donc, ni plus ni moins,

il nous paraît indispensable que la France agisse, dès ce projet de loi de finances pour 2019, et montre ainsi l'exemple à ses voisins

sur lequel l'opinion publique attend, clairement, les politiques, notamment les parlementaires. On parle beaucoup de fiscalité ; celle-ci touche parfois des gens très modestes, des gens qui travaillent. Une partie de

l'OCDE a publié un rapport dans lequel cet effet d'aubaine est clairement identifié : « Idéalement, seule la " RD marginale " devrait être subventionnée- celle que l'entreprise ne ferait pas sans la subvention -, mais cette part de la RD est impossible à isoler du reste. d'aubaine accroît le coût de la mesure pour l'État et en dilue l'impact. Afin de limiter cela, une solution consiste à asseoir la réduction d'impôt non pas sur le volume, mais sur la variation de la dépense de RD par rapport à

Premièrement, il vise à limiter le taux du CIR accordé aux grands groupes. Ce taux est actuellement fixé à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et à 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.